Nous verrons comment se dérouleront nos débats au cours de cette matinée. Interrogeons-nous du moins sur le sens politique de ce qui s'est passé hier, sur le sens politique de l'absence de la majorité sénatoriale sur ce texte, qui est pourtant son texte,

en étendant aux cas de franchissement des frontières internes la possibilité de relever les empreintes digitales. Cette possibilité est aujourd'hui limitée aux étrangers en situation irrégulière contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers à l'espace Schengen. à l'espace Schengen. Or, le refus d'entrée visant un étranger se situant hors du territoire national, il apparaît dès lors difficile de justifier l'enregistrement de ses données biométriques, d'autant qu'il peut toujours faire l'objet d'un enregistrement dans une application de police ajustée spécifiquement aux zones d'attente et dédiée à la gestion des étrangers non admis. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir un enregistrement complémentaire dans l'AGDREF, Cette mesure irait même à l'encontre de l'objectif gouvernemental, l'étranger ayant vocation à retourner rapidement dans son pays de départ.

plusieurs parquets se sont ouverts du problème auprès de votre serviteur ; ils lui ont expliqué qu'il serait particulièrement utile aux forces de police déployées à la frontière terrestre de pouvoir mieux contrôler les personnes qui y font l'objet de procédures dites de « refus d'entrée

de l'ordre la possibilité de relever systématiquement les empreintes digitales aux fins de vérification d'identité et de consultation du fichier des personnes recherchées, dans le cadre, j'y insiste, des procédures de non-admission menées depuis le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures Dès lors qu'en stricte conformité avec le code frontières Schengen le rétablissement des contrôles d'entrée et de sortie permet des vérifications approfondies, qui incluent des vérifications des empreintes digitales et des consultations des fichiers, des fichiers, les dispositions de cet article ne nous paraissent pas utiles. En effet, les personnes placées en zone d'attente à la suite des refus d'entrée sont réputées,

nous considérons que la possibilité de bénéficier d'un regroupement familial est une condition indispensable pour une bonne intégration dans notre pays, dès lors que la personne étrangère en situation régulière doit vivre et s'installer dans notre pays. Nous ne comprenons donc pas cette disposition, qui est à l'évidence contraire aux conditions d'une bonne intégration. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article. présenter l'amendement n° 422. Le Gouvernement a déposé un amendement de suppression de cet article, introduit par la commission des lois, qui durcit les conditions du regroupement familial.

familial. La directive du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial prévoit que le demandeur doit pouvoir être rejoint par sa famille au plus tard après deux ans de séjour régulier. L'administration dispose quant à elle d'un délai de six mois pour instruire un dossier de regroupement familial. Dans ces conditions, le demandeur doit pouvoir être admis à déposer sa demande

L'article 8 de cette directive indique que « les États membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur territoire pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans, avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille ». Introduire une condition de résidence préalable de vingt-quatre mois excède donc les marges d'appréciation laissées à la discrétion des États membres, sans qu'une justification suffisante soit avancée.

la conformité de cet article au droit européen, l'article 8 de la directive du 23 septembre 2003 dispose que « les États membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur territoire pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans, avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille ». Cette condition de séjour

la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que cette condition de séjour de deux ans « n'a pas pour effet d'empêcher tout regroupement familial, mais maintient au profit des États membres une marge d'appréciation limitée en leur permettant de s'assurer que le regroupement familial aura lieu dans de bonnes conditions, après que le regroupant a séjourné dans l'État d'accueil pendant une période suffisamment longue pour présumer une installation stable et un pour présumer une installation stable et un certain niveau d'intégration ». L'un des enjeux de l'immigration régulière est évidemment de rechercher cette qualité d'intégration nécessaire ; nous souhaitons tous naturellement que cette dernière soit parfaitement réussie. C'est dans ces conditions que, ne souhaitant pas, je le redis,

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Meurant, pour explication de vote.

en essayant de donner un peu de hauteur à ce débat. C'est bien ! Dans l'objet de votre amendement, monsieur Meurant, vous distinguez immigration de travail et immigration de peuplement. J'ai envie de vous poser une simple question. Il y a aujourd'hui 1,8 million de Français à l'étranger, représentés par

? Il s'agit du droit à pouvoir mener une vie familiale normale dès lors que l'on est sur le sol de la République. C'est une condition de l'intégration. Soit c'est du cynisme, soit c'est à se demander, monsieur Meurant, si vous avez vraiment compris ce que vous nous avez proposé.

de droit beaucoup plus strictes et beaucoup plus respectées. Si nous en sommes à nous poser des questions sur le regroupement familial, sur l'immigration, c'est que nous sommes dans l'incapacité d'avoir une politique migratoire, au sens large, concrète et réelle. Nous sommes dans la soumission

Le scrutin est ouvert.

J'ajoute qu'il est totalement irresponsable, les relations bilatérales de la France avec tous les pays du monde, et, en particulier avec les pays d'Afrique francophone, étant

aussi parler d'autres pays avec lesquels nous avons besoin de coopération en matière de sécurité. Il serait tout aussi irresponsable de conditionner tous nos efforts diplomatiques à la délivrance des laissez-passer consulaires. L'égalité entre les citoyens du monde exige que leurs demandes de

453. Il arrive, et nous sommes en train de le vérifier, que l'on présente la même proposition avec des argumentations extrêmement différentes. Je suis en désaccord complet avec tout ce que vient d'expliquer l'orateur précédent. Je crois qu'il est absolument nécessaire et rationnel, si l'on veut avoir une politique de maîtrise des flux migratoires, ce qui est vital pour notre pays et pour l'Europe, d'utiliser les moyens nécessaires, dans les rapports de souveraineté, pour obtenir des pays d'origine des flux migratoires qu'ils assument leurs responsabilités en reprenant leurs ressortissants qui ont été légalement évincés du territoire français. Cela est particulièrement vrai pour les pays avec lesquels nous avons des liens de proximité et de solidarité, mais, qui, sur ce plan, pour des raisons sociales que nous pouvons entendre, s'avèrent non coopératifs, dans des conditions directement contraires aux intérêts de la France.

Il peut se produire qu'une commission adopte ce que l'on nomme habituellement un amendement d'appel et, du coup, en fasse un article de loi. Mais honnêtement, il ne nous paraît pas du tout rationnel

S'il est vrai que l'efficacité des mesures d'éloignement est une question centrale, nous partageons les

convient, que l'efficacité de notre politique migratoire passe d'abord, en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, par l'obtention de laissez-passer consulaires des pays sources. Je ne vais pas citer

à celle de laissez-passer consulaires, c'est-à-dire au fait que ces pays acceptent de reprendre sur leur territoire des ressortissants en situation irrégulière sur le nôtre. Il ne s'agit rien de plus. Par ailleurs, cet article est conforme aux dispositions réglementaires et aux conventions internationales. Je rappelle à cet égard que l'Europe est en train de travailler

du Gouvernement ? La commission des lois a adopté cet article qui permet de refuser un visa de long séjour à un étranger au motif que l'État dont ce dernier a la nationalité n'est pas suffisamment coopératif pour réadmettre ses ressortissants faisant l'objet en France d'un mesure d'éloignement. Il est vrai que l'obtention de laissez-passer consulaires est un déterminant de l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière, et, comme vous le savez, le Gouvernement est pleinement mobilisé à cet effet. Je peux en attester personnellement pour avoir travaillé

me suis rendue. Cependant, le taux de délivrance des laissez-passer consulaires ne saurait justifier les dispositions de l'article 11 A selon lesquelles l'autorité administrative pourrait décider pourrait décider de refuser ou non un visa de long séjour à un particulier sans autre critère que sa nationalité. Ces problèmes ô combien essentiels ne sauraient se régler dans le cadre d'un

À cet égard, le Gouvernement conduit une action résolue pour accroître la délivrance par les pays d'origine de ces documents. Cela passe par l'action diplomatique menée non seulement par le Président de la République et le Gouvernement, mais aussi par l'ambassadeur des migrations, qui intervient auprès des pays d'origine, ainsi que par la mise en place au ministère de l'intérieur d'une

le nombre d'éloignements a augmenté de 14 % par rapport à 2016. C'est encore insuffisant, nous le savons, mais je voulais le signaler. Sur les quatre premiers mois de la

L'attribution d'un visa, c'est une prérogative de souveraineté que la République française exerce, avec un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner que celle-ci puisse décider tout à fait librement de sa pratique en la matière. J'en viens, La disposition adoptée par la commission des lois et que plusieurs amendements tendent à supprimer est respectueuse des prérogatives diplomatiques du gouvernement français. Elle ne lui fait aucune injonction.

qu'il viole les dispositions d'un accord passé avec elle, soit qu'il fasse preuve de mauvaise volonté pour la délivrance, par exemple, de certificats consulaires pour ses ressortissants en instance d'éloignement et que nous ne pouvons pas éloigner tant que nous n'avons pas la confirmation de leur identité et de leur nationalité. C'est l'objet même de ces certificats consulaires. Il ne faudrait donc pas faire à la disposition adoptée par la commission des lois un excès d'indignité. Elle n'est pas frustratoire de droits qu'exerceraient des étrangers à l'égard de la République

Quand le ministre de l'intérieur va négocier avec un État étranger pour que celui-ci délivre plus facilement des certificats consulaires, il se prévaut de la volonté expresse du Président de la République en ce sens. Eh bien, désormais, si nous gardons la disposition adoptée par la commission des lois, il pourra se prévaloir aussi de la volonté expresse de la représentation nationale ! Nous donnons ainsi plus de force au ministre de l'intérieur pour ces négociations. Et c'est, de mon point de vue, une très bonne chose pour faire progresser la maîtrise des flux migratoires sans frustrer aucun droit d'aucune personne, d'aucun État ni du Gouvernement

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

Benbassa, sur l'article. Le présent article 11 comporte deux mesures particulièrement problématiques. Il prévoit, tout d'abord, qu'un étranger qui a déposé une demande d'asile et qui souhaite demander un autre titre de séjour doit effectuer cette seconde démarche cette seconde démarche en parallèle de la première. Il précise, ensuite, que, en cas de rejet de la demande d'asile et de la demande de titre de séjour, la délivrance d'une obligation de quitter le territoire français est systématique.

afin d'appréhender la situation des exilés femmes et LGBT. Les associations de défense des droits des gays ont notamment tenu à ce que nous fassions cas des dérives que le présent article pourrait entraîner à l'encontre des personnes issues de ces minorités. Par exemple, une personne homosexuelle séropositive qui n'aurait pas été bien informée sur la nécessité de formuler ses deux demandes parallèlement et qui se serait vu déboutée de sa demande d'asile, n'ayant pu « prouver » son homosexualité, se verrait signifier une obligation de que sa condition sanitaire aurait pu lui permettre d'être éligible à un titre de séjour pour motif de santé. Ces mesures ont pour effet de limiter de manière significative le droit des exilés à bénéficier d'un titre de séjour. limite également la possibilité pour les requérants de fonder sereinement leurs dossiers. Ces éléments sont particulièrement préoccupants, notamment pour les cas que nous venons de soulever. Nous ne pouvons accepter la précarisation de populations déjà si fragiles

Je ne les excuse pas, mais je justifie leur absence. Je trouve en effet que la réponse qu'on apporte aujourd'hui à cette problématique extrêmement grave qu'est l'immigration est bien en deçà de ce que nous devrions faire.

que 3,5 millions de réfugiés sont basés en Turquie et qu'ils y restent par la grâce d'un accord de dupes avec ce pays, lequel peut d'ailleurs très bien ouvrir ses vannes à la première occasion ce sont surtout- et ce n'est pas moi qui le dis -20 à 25 millions de migrants potentiels, qui se pressent en Afrique, en bordure de l'Europe. M. le ministre

parce qu'il y va de notre responsabilité vis-à-vis de nos enfants ! Et je pense que c'est une lourde responsabilité

inutiles, inefficaces et indignes. Ce n'est pas une réponse, mais nous en sommes là ! Donc, nous poursuivons la discussion en nous concentrant sur des amendements qui essaient de limiter les dégâts

sur chaque amendement et sur chaque article, mais êtes-vous sûrs de pouvoir voter, tel que vous le faites, pour vos collègues absents ? Car s'ils ne sont pas là, M. Pemezec l'a dit, c'est justement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce texte.

de la commission, monsieur le rapporteur,

n° 264 rectifié, car son adoption conduirait à restreindre l'application de l'interdiction de retour aux seuls cas où elle est systématique, sous réserve de circonstances particulières.

de la commission, monsieur le rapporteur,

est en mesure d'apprécier.

le président du tribunal administratif devant pour sa part statuer dans les 72 heures après sa saisine. L'objectif du législateur était de permettre à l'autorité administrative de régler la situation d'une personne étrangère détenue avant sa sortie de détention, afin d'éviter le placement en rétention à l'issue de sa libération, ce qui correspondait à la pratique suivie avant l'entrée en vigueur de la loi de 2016. Cette disposition de la loi du 7 mars 2016 a cependant été récemment déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel

Le Conseil a notamment retenu que l'étranger disposait d'un délai trop bref, 5 jours au maximum, quelle que soit la durée de la détention, pour exposer au juge ses arguments et réunir les preuves au soutien de ceux-ci. Le Conseil a également pris en considération le fait que l'administration devrait, lorsque la durée de la détention le lui permet, procéder à la notification de l'OQTF suffisamment tôt au cours de l'incarcération, afin de laisser plus de temps à la procédure contentieuse. En conséquence, le Conseil a censuré cette disposition en ce qu'elle fixait les délais impartis à l'étranger détenu pour former un recours et au juge

En premier lieu, il ne sera plus recouru systématiquement à la procédure contentieuse accélérée, mais uniquement En premier lieu, il ne sera plus recouru systématiquement à la procédure contentieuse accélérée, mais uniquement en tant que de besoin. En effet, l'objectif de la loi de 2016 était de régler la situation d'une personne détenue, je le rappelle, avant sa sortie de détention. En conséquence, c'est seulement lorsqu'il apparaîtra que l'étranger détenu va être libéré avant que le juge statue sur l'OQTF que le basculement vers la procédure accélérée sera possible. Quand le président du tribunal administratif sera informé que la levée d'écrou va intervenir avant l'expiration du délai de jugement prévisible, il disposera alors de 144 heures, soit 6 jours pour statuer. Ainsi, l'étranger disposera désormais de 8 jours, correspondant aux 48 heures du délai de recours en cas de refus du délai de départ volontaire et aux 144 heures allouées au juge pour se prononcer,

Il convient au demeurant de souligner que cette hypothèse de 8 jours constitue un cas extrême, lorsque l'OQTF est notifiée dans les derniers jours de la détention. Dans les autres cas, le délai ouvert à l'étranger sera nécessairement plus long.

Si je partage, bien entendu, l'objectif du législateur d'éviter de faire se succéder une période de rétention à une période de détention, ce qui implique que l'administration procède aux diligences nécessaires en notifiant les OQTF suffisamment tôt en amont de la levée d'écrou, je ne peux que contester la rédaction proposée par le Gouvernement dans son amendement n° 146. En effet, cet amendement, s'il était adopté, ne réglerait rien et ferait toujours encourir un risque d'inconstitutionnalité des dispositions qu'il contient. Le Gouvernement s'attache à donner davantage de temps au juge pour statuer- 144 heures, soit 6 jours -, mais semble peu regardant quant au délai de recours accordé au détenu pour contester l'OQTF notifiée en détention. l'amendement n° 353, nous proposons une solution simple, respectueuse du droit à un recours effectif et qui a le mérite d'unifier les procédures, en s'alignant sur les délais prévus au I de l'article L.512-1 du CESEDA, à savoir un délai de recours de 15 jours pour contester les OQTF et un délai de 6 semaines laissé au juge pour statuer. statuer. Si toutefois l'administration n'a pas notifié suffisamment tôt l'OQTF et que la date de la levée d'écrou doit intervenir avant la fin du délai de recours, le détenu pourra bénéficier du reliquat du délai restant à la levée d'écrou pour former son recours, sans qu'il soit pour autant « perdu dans la nature ». Bien Bien entendu, il sera alors placé sous le régime du III de l'article L. 512-1 précité et soumis aux délais et procédures applicables aux personnes retenues ou assignées à résidence. Concrètement, le juge devra alors statuer dans les 72 heures afin d'éviter que ne se prolonge la période de rétention, si elle n'a pu être évitée en raison d'une notification trop tardive de l'OQTF.

et ses droits à demander l'assistance d'un interprète et d'un avocat. C'est essentiel, puisque les détenus ne peuvent pas conserver en cellule de document où figure le motif d'écrou, ce qui est pourtant le cas de la quasi-totalité des OQTF.

la ministre, mes chers collègues, l'article 14 est des plus contradictoires. Il prévoit en effet la possibilité d'assigner à résidence les étrangers qui font l'objet d'une OQTF avec délai de départ volontaire. Mes chers collègues, j'ai beau chercher la cohérence de cet article, je ne la trouve pas ! D'un côté, il est prévu de faire confiance à l'étranger s'étant vu signifier une OQTF, en lui laissant un délai de départ volontaire ; de l'autre, nous lui demandons de rester dans un périmètre qui aura été choisi par l'administration compétente. Ainsi, deux points me frappent à la lecture de cet article. En premier lieu, la décision d'assigner à résidence est prise sans considération individuelle, sans tenir compte des situations personnelles et médicales des exilés concernés. En second lieu, une logique insidieuse se glisse une fois de plus au sein de ce de laquelle les exilés sont des criminels prêts à prendre la fuite. Jusqu'à présent, ces mesures n'étaient appliquées qu'aux personnes suspectées de terrorisme, dans le cadre de l'état d'urgence. Avec cet article, elles seraient généralisées à tous les exilés. Quoi que fasse le Gouvernement, pour l'heure et en l'état du droit, être sans papiers n'est pas une infraction à la loi. Cessons de traiter les exilés comme des tenants du grand banditisme et laissons à ceux qui se sont vu signifier une obligation de quitter le territoire français la possibilité de rendre cette demande de l'administration effective

s'agit de supprimer la possibilité d'assigner à résidence un étranger qui fait l'objet d'une OQTF avec délai de départ volontaire.

Tout à l'heure, il a été rappelé que, sur les 85 000 mesures prononcées en 2017, seules 15 000 avaient été exécutées,

C'est pourquoi le texte prévoit de désigner aux personnes concernées un lieu de résidence, ce qui permettra d'assurer un meilleur suivi et de les localiser, si elles ne répondent pas aux convocations de l'administration.

Si l'on propose qu'une OQTF soit applicable avec un délai de départ volontaire, cela signifie que l'on considère que la personne doit partir,

le cas des étrangers non européens bénéficiant d'un titre de séjour valide en France, puisqu'il a été délivré par un autre État membre de l'Union européenne. Nous notons une contradiction fondamentale du point de vue du droit au sein du traité de Schengen lui-même, puisque ce texte prévoit explicitement l'élargissement de cette interdiction. En effet, l'espace Schengen est censé organiser la libre circulation des travailleurs disposant de titres de séjour tout en prévoyant des dérogations à ce principe. Ce qui nous pose le plus de problèmes, c'est la discrimination établie sur notre territoire entre deux étrangers disposant chacun d'un titre de séjour, selon que celui-ci est accordé en France ou ailleurs dans l'Union européenne.

faisant l'objet d'une remise à un autre État membre. Il s'agit ainsi de garantir l'effet utile des « remises Schengen » et d'éviter qu'une personne éloignée vers un autre pays de l'espace Schengen ne revienne rapidement sur le territoire français, en bénéficiant de la libre circulation.

La commission des lois a en effet généralisé et systématisé le prononcé des peines d'interdiction du territoire, qui entraînent de plein droit la reconduite du condamné à la frontière. Celles-ci seront désormais prévues pour toute infraction

bien définie, qui a juridiquement pour objet de parer à une menace : elle a un caractère préventif et non répressif. Elle constitue non pas une sanction, mais « une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics l'autorité administrative doit se fonder sur l'ensemble du comportement de l'étranger, sans même avoir besoin de fonder sa décision sur une inscription à un quelconque fichier ou une peine antérieure de prison. La sanction ne saurait donc être automatique sans encourir la censure du Conseil constitutionnel.

en situation irrégulière et 80 étrangers en situation régulière ont fait l'objet d'une mesure administrative d'expulsion ou d'éloignement, que celle-ci soit exécutée ou en cours d'exécution.

Le recours à des moyens de télécommunications audiovisuelles pour la tenue des commissions départementales d'expulsion est actuellement seulement prévu pour le cas spécifique de Mayotte. Toutefois, Toutefois, le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement, car, en dehors du fait que la nécessité d'une telle disposition n'est pas établie, la rédaction proposée manque de précision et ne prévoit pas les garanties qui doivent entourer le recours à cette technique pour assurer le bon déroulement de la procédure de consultation de la commission. Dès lors, son usage dans ce cadre soulèverait plusieurs difficultés et ne manquerait pas d'être sanctionné par le juge. Pour ces motifs, le Gouvernement émet un avis défavorable

ont ainsi connaissance des mesures par lesquelles les autorités administratives prononcent des éloignements du territoire. Ainsi peuvent-ils mettre fin au versement des prestations ou aides allouées ou prendre toutes les décisions tirant les conséquences de ces informations, dans le respect des réglementations propres à chacune de ces prestations. Afin de rendre plus efficient l'usage des informations relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement en vue de mettre fin aux versements des prestations ou aides allouées, le Gouvernement souhaite par ailleurs favoriser l'échange des informations avec les organismes précités. Il n'est en revanche ni nécessaire ni pertinent d'insérer une disposition générale dans le CESEDA, qui n'a pas vocation à contenir les règles d'attribution des prestations sociales et qui ne permettrait pas de prendre en compte les caractéristiques propres à chacune de ces prestations.

Comme l'a dit Mme la ministre, il nous faut assurer la coordination entre les organismes publics chargés de l'un et de l'autre- je n'ai aucun mal à croire qu'elle soit encore améliorable -, mais confier à l'autorité de police,

Gontard, sur l'article. L'article 15 , qui a été introduit par la commission des lois du Sénat, va, une fois n'est pas coutume, dans le bon sens. Il interdit le placement en rétention des mineurs isolés. En effet, comme cela est indiqué dans le rapport, cette interdiction résulte en France d'une combinaison peu lisible de plusieurs dispositions législatives. Cette combinaison est si peu lisible que, selon une note du Défenseur des droits en date du 25 mai dernier, les placements d'enfants augmentent de façon soutenue en métropole : en 2017, quelque 305 enfants ont été placés en centre de rétention en métropole, soit sept fois plus qu'en 2013. À Mayotte, 4 325 mineurs ont été enfermés en 2016, contre 2 493 en 2017. Parmi eux, des enfants seuls sont rattachés de manière arbitraire et illégale à un adulte, également en voie d'éloignement, sans que celui-ci exerce sur eux une autorité parentale. Il s'agit de rendre possible leur rétention. Le rapport de la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, publié il y a quelques jours, le 6 juin, sur la situation des mineurs à la frontière franco-italienne est également éloquent sur ce genre de dérapages parfaitement intolérables Les mineurs isolés représentent près d'un tiers des personnes non admises à la frontière franco-italienne (10 434 mineurs ont fait l'objet d'une procédure d'un refus d'entrée à Menton entre janvier et septembre 2017 selon les chiffres fournis par la direction départementale de la police aux frontières), ils ne font pour autant pas l'objet d'un traitement très différent de celui des adultes. » Selon la police aux frontières, les mineurs voyageant à plusieurs ou accompagnés d'adultes de la même nationalité ou parlant la même langue sont considérés comme « faisant famille ». Or, comme le recommande le Comité européen pour la prévention de la torture, « les enfants non accompagnés ou séparés qui sont privés de liberté doivent obtenir rapidement et gratuitement l'accès à une assistance juridique, ou à une autre assistance appropriée, y compris la désignation d'un tuteur ou d'un représentant légal, qui les tient informés de leur situation juridique et protège effectivement leurs intérêts ». Si cet article va dans le bon sens, il convient d'être vigilant sur l'article réitère une interdiction qui est censée déjà exister, mais qui est enfreinte au quotidien par les autorités publiques. Ensuite, l'interdiction posée est limitée, hélas, à une catégorie de mineurs, les mineurs isolés, quand ceux-ci ne sont pas rattachés à une famille fictive. Or, nous en avons déjà parlé et nous le verrons dans la suite du débat lors des interventions de mes collègues, il est de notre responsabilité aujourd'hui d'interdire la rétention pour tous les mineurs, sans exception, y compris ceux qui sont accompagnés de leur famille. La parole est à M. Jean-Yves Leconte,

et a signalé l'atteinte à l'intégrité psychique que représente une incarcération pour des mineurs, quelle que soit leur situation. La Cour européenne des droits de l'homme, en 2016, a condamné six fois la France sur cette question. L'encadrement proposé par la commission des lois, s'il

Disons les choses clairement : votre proposition revient à empêcher l'éloignement de tout mineur en situation irrégulière.

général des lieux de privation de liberté. J'en viens à l'amendement n° 25. Comme je l'ai dit mardi, le Sénat s'honorerait en adoptant un dispositif de protection des mineurs étrangers. Je me permets d'insister de nouveau aujourd'hui sur cette question. Les mineurs ne sont pas des migrants. Ce sont des enfants, et ce jusqu'à leurs 18 ans et une seconde. Nous avons vu les tensions que font naître les questions éminemment importantes de la protection des femmes qui sont persécutées dans leur pays,

du respect de nos principes fondamentaux et des normes supranationales. Nous avons déjà dénoncé toutes les atteintes à ces principes, mais il s'agit d'abord et avant tout d'une question d'humanité.

La protection de l'intérêt supérieur de l'enfant est une des lignes directrices qui ont guidé notre positionnement sur ce texte, comme auparavant lors de l'examen de la proposition de loi Warsmann. Nous saluons donc la proposition du rapporteur d'inscrire dans la loi l'interdiction de placer en centre de rétention administrative des mineurs non accompagnés. Monsieur le rapporteur, c'est un premier pas ! Mais la situation la plus préoccupante aujourd'hui est celle des mineurs accompagnant leurs parents, eux aussi placés en centre de rétention administrative. Ces placements se sont intensifiés au cours des dernières années. 275 enfants ont été placés en centre de rétention en 2017, soit autant que les quatre années précédentes, de 2012 à 2015.

C'est vrai, mais de notre point de vue, l'assignation à résidence devrait toujours être préférée au placement en centre de rétention administrative, s'agissant de mineurs, accompagnés ou non. Tel est l'objet de cet amendement.

Arnell. Cet amendement de repli vise à contraindre l'autorité préfectorale prononçant une décision de placement en centre de rétention administrative à spécialement motiver sa décision lorsqu'elle concerne le placement de mineurs. Ces motivations visent à prouver l'examen scrupuleux de la vulnérabilité personnelle de l'enfant, ainsi que la prise de dispositions particulières relativement à sa minorité. cette disposition devrait contraindre les préfectures à ne recourir au placement d'enfants en centre de rétention administrative que de manière très exceptionnelle.

peut-on ou non placer un enfant mineur en rétention, qu'il soit seul ou accompagnant de sa famille ? Ni le texte d'origine du Gouvernement ni les débats à l'Assemblée nationale n'ont apporté, de quelque manière que ce soit, de réponse à cette question difficile, car elle est difficile.

sensibilité de ce sujet. La rétention familiale, c'est-à-dire la rétention des parents avec leurs enfants mineurs, fait l'objet de débats. Nous l'avions d'ailleurs constaté lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, sur ce sujet dont, encore une fois, je comprends l'extrême sensibilité, je tiens à apporter quelques explications et précisions. Tout d'abord, je le rappelle, la rétention familiale est une procédure exceptionnelle, qui fait l'objet d'un encadrement strict. Elle est exceptionnelle, car, même si le droit européen l'autorise, nous devons nous assurer que l'intérêt de l'enfant prime et nous devons protéger les mineurs contre tout abus de placement en rétention. C'est ce que nous faisons. nous faisons. En 2017, les mineurs accompagnants en rétention ne représentaient que 1,17 % de l'ensemble des personnes placées en rétention en métropole. Ensuite, il s'agit d'une procédure strictement encadrée. Elle intervient lorsque la famille s'est déjà soustraite à une procédure d'éloignement, autrement dit, lorsque la famille, placée en assignation à résidence, a a fui le domicile ou a placé ses enfants ailleurs pour faire échec à la mesure d'éloignement. Je répète qu'on ne peut pas faire appliquer la mesure d'éloignement si les enfants ne sont pas présents. si le placement en rétention de l'étranger dans les 48 heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne de certaines contraintes liées à la nécessité de leur transfert. En outre, je précise que notre droit permet que seuls les parents soient placés en rétention. Les enfants mineurs, pendant ce temps, peuvent être placés en famille d'accueil. Toutes les familles peuvent avoir recours à cette possibilité.

que nous faisons le maximum pour que la durée de la rétention soit la plus courte possible. Le 12 juillet 2016, la Cour européenne que la durée de rétention des familles doit être la plus courte possible, avait estimé qu'une durée de 18 jours était disproportionnée par rapport au but recherché et constituait en l'espèce

Face à un refus d'embarquer, il faut prévoir l'organisation d'un nouveau vol, ce qui prend inévitablement quelques jours.

Strictement encadrée, cette procédure est donc nécessaire et existe aussi chez nos voisins européens. La rétention des mineurs accompagnant leurs parents, pardon des enfants mineurs- un certain nombre d'entre vous tiennent à ce mot, ce que je comprends doit rester une possibilité afin de garantir la crédibilité de notre politique d'éloignement. La Commission européenne a d'ailleurs, dans sa recommandation du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs, expressément recommandé aux États membres de l'Union européenne de ne pas interdire le placement en rétention des familles, sous peine de priver d'efficacité les politiques d'éloignement. Toute décision contraire priverait d'effet utile la directive Retour et placerait la France dans un cadre qui ne respecterait pas ses obligations communautaires.

Conformément au droit français, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un enfant mineur n'est possible que dans un lieu bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.

certains s'étant simplement rendus coupables d'infractions au droit des étrangers et d'autres, plus dangereux, attendant d'être expulsés en raison de la menace pour l'ordre public que représente leur présence sur le territoire national. Afin Afin d'assurer la sécurité des personnes les plus vulnérables placées dans ces centres, mais aussi celle du personnel, nous proposons que

? Monsieur Arnell, vos préoccupations sont, bien sûr, tout à fait pertinentes. La sécurité des personnes doit être garantie dans les centres de rétention administrative. Et elle l'est,

dont il a la charge. Il incombe à ce dernier, dans ce cadre, de prendre toutes les mesures utiles et proportionnées pour assurer la sécurité de tous, le cas échéant en séparant déjà ceux qui sont retenus dans les CRA.

au mieux une fausse bonne idée, pouvant même entraîner des dérives. Certes, ni le Gouvernement ni les députés En Marche n'ont mis fin à la rétention des familles avec mineurs, la loi permettant, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, de les retenir 3 mois dans des lieux totalement inadaptés. Mais inscrire une durée maximale de 5 jours pour la rétention des familles n'apporte pas de protection supplémentaire aux enfants ; cela vient au contraire banaliser cette pratique et, indirectement, donner l'autorisation d'enfermer des familles pendant 5 jours. Or le traumatisme que représente l'enfermement pour un enfant, qui intervient souvent après un périple épuisant pour arriver en France, ne dépend pas de la durée de rétention. L'UNICEF relève d'ailleurs, quelle que soit cette durée, de graves conséquences sur la santé physique et psychique des enfants enfermés. De nombreuses études récentes, notamment anglo-saxonnes, ont en effet démontré que l'enfermement, même pour une brève période, entraîne chez l'enfant de multiples troubles tels que ceux qui sont observés lors d'un état de stress post-traumatique : anxiété, dépression, troubles du sommeil, importante perte de poids, refus de s'alimenter, troubles du langage et du développement. Ainsi, et comme le rappelle la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 12 juillet 2016, « il convient de garder à l'esprit que la situation d'extrême vulnérabilité de l'enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d'étranger en en séjour illégal ». Les directives européennes encadrant la rétention des étrangers considèrent à ce titre que les mineurs, qu'ils soient ou non accompagnés, comptent parmi les populations vulnérables nécessitant l'attention particulière des autorités. En effet, les enfants ont des besoins spécifiques dus notamment à leur âge et à leur état de dépendance. Or les conditions d'organisation des centres de rétention ne peuvent qu'avoir un effet délétère sur les enfants. Quand on légifère, il faut penser aux conditions réelles de l'application de la loi. Par ailleurs, dans une récente décision de juin 2017 concernant deux fillettes maintenues en zone d'attente, le Défenseur des droits a pu mettre en lumière les atteintes au droit et à l'intérêt de ces deux enfants, ce qui plaide ainsi en faveur de plusieurs modifications législatives. Comme je viens de le souligner et tel que notre débat l'a mis en exergue, cet article ne va pas dans le bon sens, tout au contraire. Assassi, sur l'article. L'article 15 vient alimenter un droit interne inadapté aux normes supranationales, en introduisant désormais dans la loi l'enfermement des familles avec enfants. La préservation de l'unité familiale fait partie intégrante de l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsqu'un enfant est avec ses parents, l'administration ne doit pas les séparer. L'argument, souvent avancé sur différentes travées, consistant à dire que certains adultes, accompagnés ou non d'enfants, doivent être enfermés en raison du danger ou de la menace qu'ils représenteraient, est absurde et ne peut être entendu. Mes chers collègues, un individu représentant un danger ou une menace pour n'importe qui l'est d'abord pour les enfants qui l'accompagnent. Dans ce cas, il va sans dire que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être recherché lorsque la protection du parent est défaillante : il doit relever des services départementaux compétents de l'aide sociale à l'enfance. Selon la loi en vigueur, tout placement d'une famille en rétention implique que celle-ci a, avant son enfermement, enfreint les conditions de son assignation à résidence ou bien a pris la fuite à l'occasion d'une mesure d'éloignement, la rétention étant alors présentée comme le « dernier recours ». Pour sa part, la Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande que l'enfermement d'enfants soit interdit dans les centres de rétention administrative », précisant que « seule la mesure d'assignation à résidence [peut] être mise en oeuvre à l'égard des familles accompagnées d'enfants ». Dans la pratique, le placement de familles en rétention est souvent moins une exception qu'un mode de fonctionnement pour certaines préfectures. Les préfectures du Doubs et de la Moselle totalisent 51 % des placements de familles réalisés en 2016. À l'inverse, le centre de rétention de Lille-Lesquin, pourtant habilité à accueillir des familles, y a renoncé depuis la condamnation de la France par la CEDH en 2012.

Benbassa, sur l'article. Peut-on se féliciter que ce projet de loi vienne limiter dans le temps la présence d'enfants dans ces centres, alors même qu'il prévoit le rallongement de la durée de détention pour les autres personnes retenues et que la majorité présidentielle, à l'Assemblée nationale, s'est refusée à proscrire leur présence en CRA ? Non, bien évidemment ! D'une part, déterminer une durée de rétention pour les mineurs exilés dans la loi, c'est légitimer la présence des familles en CRA. D'autre part, la simple idée qu'un enfant puisse se trouver en ces lieux dépasse toute humanité et tout entendement raisonnable. Ce sont de véritables lieux d'enfermement, gérés, je vous le rappelle, par la police. Des enfants, quelle que soit la situation administrative de leurs parents, n'ont rien à y faire. C'est à la fois l'avis de Mme Hazan, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, de M. Toubon, Défenseur des droits, mais aussi de nos concitoyens. En atteste la pétition à ce sujet de l'UNICEF, qui a recueilli plus de 100 000 signatures. Dans son rapport, la Contrôleur général détaille avec horreur l'impact des CRA sur le développement infantile, ma collègue Laurence Cohen : troubles anxieux et dépressifs, perte de poids, sommeil perturbé, troubles du langage et du développement psychique. Avec ces données sanitaires, comment le Gouvernement peut-il refuser d'interdire la présence juvénile au sein des centres de rétention ? Après pas moins de six condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour rétention administrative d'enfants, il est urgent d'y mettre

L'objet de cet amendement est de supprimer l'article 15 introduit par la commission des lois

droits de l'homme, les enfants étaient maintenus en rétention pour une durée supérieure à 2 semaines.

Madame la ministre, la commission des lois est coopérative. Elle a conscience des enjeux que représente l'éloignement des étrangers, y compris des étrangers qui vivent en France, en famille, de manière irrégulière. Aussi bien avons-nous permis, par la disposition adoptée en commission, que ces familles soient retenues jusqu'à 5 jours en centre de rétention. Mais la réponse que vous nous apportez ne peut nous satisfaire,

dans la position de devoir faire la balance entre deux aspects qui paraissent disproportionnés : l'éloignement des familles, nécessaire quand elles sont en situation irrégulière, mais aussi notre devoir d'humanité à l'égard des enfants. été très sensible à ce qui a été dit. Nous partageons tous cette idée qu'il n'est pas digne de notre République et de notre État de droit de prolonger le séjour d'enfants qui sont, par hypothèse, innocents, même quand ils sont instrumentalisés

ministre, je vous le dis tout net, le Sénat ne peut accéder à votre demande pressante d'annuler cette disposition, somme toute bien modérée.

montre d'humanité sans allonger exagérément le propos. Il me semble simplement que la position retenue par la commission, que je n'avais pas suivie pendant le débat de commission, manque une partie de son objectif. En effet, comme l'a dit le président Bas à plusieurs reprises,

et non d'une durée courante, la commission serait plus conforme à son objectif en adoptant une durée de 10 ou 12 jours. C'est la raison pour laquelle je ne voterai pas son texte. Je vais mettre aux voix

Or, aujourd'hui, nous en venons à considérer la restriction à 5 jours, proposée par M. le rapporteur et adoptée en commission, comme un progrès pour les droits des enfants, au regard de ce que propose le Gouvernement- et c'est vrai !

de la conscience socialiste. En effet, la dernière fois que j'ai vu des membres de votre famille politique défendre l'interdiction de la rétention des enfants, c'était le 14 mars 2012,

Ce silence est devenu particulièrement assourdissant lorsque nous avons examiné les textes relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, en 2015 et en 2016. Le temps a passé,